Par ailleurs, dans l'enquête que nous avons menée auprès d'un échantillon représentatif de maires français, 90 % des élus sondés estimaient que cette instance devait être obligatoire.

pour pouvoir rendre sa création obligatoire dans l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Chacun peut s'étonner que la commission soutienne une proposition visant à rendre obligatoire la création d'une institution, mais cela me semble aller dans le sens que nous défendons depuis le début, à savoir redonner aux maires

que, dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, on décide de la création de la conférence des maires. Dès lors que le pacte de gouvernance est facultatif,

là où les maires pourraient être exclus de la gouvernance, là où ils seraient empêchés de donner leur avis sur le projet de territoire, là où ils ne seraient pas associés à la vie de l'intercommunalité,

Et, pendant ce temps-là, on ne s'interroge pas sur les dysfonctionnements du système actuel des intercommunalités, que l'on a voulues gigantesques, où certains élus se sentent noyés, dans lesquelles les communes ne sont pas représentées

proposons une conférence des maires à caractère obligatoire. Toutefois, nous confions au pacte de gouvernance

je vous invite à vérifier que votre carte de vote est bien insérée dans votre terminal. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater les résultats du scrutin.

Dans de nombreux territoires, certains élus ont souvent fait part de leur désarroi lors de situations inverses : si certains EPCI ont déjà engagé des démarches pour mieux les associer, ce n'est pas le cas de tous. loi, le Gouvernement entend agir sur ce point. En effet, l'article 1 offre la possibilité aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines d'organiser une conférence des maires.

À mon sens, il est très important que chaque maire ait voix au chapitre : les décisions ne se prennent pas dans l'instant, elles se préparent où vous savez

plus grandes. Notre groupe maintient donc sa position sur le caractère obligatoire de cette instance, qu'il avait déjà fait adopter par le Sénat en janvier 2019, lors de l'examen de la proposition de loi socialiste visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires. Nous restons sur cette ligne.

La conférence des maires est une instance de dialogue et de coordination particulièrement utile quand tous les maires des communes membres d'un EPCI ne siègent pas en son bureau. Cet amendement vise donc à rendre sa création obligatoire dans une telle situation.

allant dans le sens de l'obligation de la création d'une conférence des maires dans chaque EPCI semble grandir. Pour ce qui nous concerne, nous retirons cet amendement au bénéfice de celui de M. Jean-Marie Mizzon, en considérant qu'une intercommunalité ne peut se construire que dans le consensus et le compromis et qu'il n'y a pas mieux que les maires pour le rechercher et l'obtenir.

a adopté un amendement qui tend à rendre la création d'une conférence des maires obligatoire dans les métropoles, mais facultative dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

la majorité qui viendra d'être désignée, ce n'est pas chose aisée. Afin d'assouplir les possibilités de faire vivre la démocratie locale, nous proposons donc de faire passer

adresser à nos territoires et à nos collègues élus locaux. Liberté, liberté, liberté ! Cessons d'invoquer Tocqueville alors que, une fois de plus, on parle d'obligation

Je me souviens que, dans cet hémicycle, lors de l'examen d'un précédent texte de réforme des collectivités locales, Jean-Pierre Chevènement, qui était sénateur et qui est, comme vous le savez, le père de l'intercommunalité, avait rappelé qu'en créant les communautés de communes,

Marie ! Ces sujets, manifestement, ne concernent pas seulement notre groupe, mais semblent être partagés par d'autres groupes et par bon nombre de nos collègues ici présents, qui ont une expérience de l'intercommunalité. Monsieur le ministre,

sentir entendue. Nous essayons de trouver un substitut à cette incapacité de penser l'intercommunalité en permettant aux petites communes d'avoir leur part de pouvoir, et donc d'information automatique devant la décision.

groupe le répète depuis le début de cette séance, je ne suis pas convaincue que rendre obligatoire la conférence des maires

n'ai pas eu l'impression d'être un plus petit adjoint que celui de la ville d'à côté. C'est le charisme, le bon sens et l'honnêteté de chacun qui fait la qualité de la gouvernance de la communauté de communes, non une loi qui obligerait à faire des choses qui ne sont que facultatives.

au charisme et à l'intelligence de chacun. Il y aura des élections municipales au printemps, les électeurs essayeront de choisir les gens les plus capables pour diriger leur commune et pour la représenter au sein des divers organismes, tels que la communauté de communes ou les quelques syndicats qui existent encore

Pour moi, c'est de défendre le plus faible. La loi peut être appréhendée de manières différentes : elle doit bien sûr servir l'intérêt général, mais il est des lois, qui prennent en compte les intérêts des plus petits. Actuellement, à l'Assemblée nationale, se trouve en discussion une loi qui porte sur une minorité ; mais cela n'en fait en rien une petite loi.

dans la discussion générale que le projet de loi que vous nous soumettez avait pour caractéristique l'esprit d'écoute,

Personne ne demande plus à voter ? ... Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater les résultats du scrutin.

: La parole est à M. Jean-Yves Roux. Cet amendement a pour objet de prévoir que le pacte de gouvernance doit préciser les modalités par lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte au sein des conseils municipaux des actions engagées en faveur de chaque commune. Il s'agit de créer un outil dont les modalités doivent être adaptées au cas par cas, procédant de la logique de renforcement de l'évaluation par la commune des actions menées par l'intercommunalité. L'objectif est également de renforcer les liens et les synergies entre conseils municipaux et EPCI, tout en rapprochant le maire des centres de décision.

vise à supprimer la disposition prévoyant que les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par le pacte de gouvernance. En effet, cet alinéa entretient une confusion entre ce qui relève de ce pacte, qui, comme son nom l'indique, est destiné à définir les modalités de gouvernance de l'intercommunalité,

de la commission ? Il nous semble que le fonctionnement et l'organisation des commissions intercommunales, comme ils procèdent de la volonté d'associer le plus largement possible l'ensemble des conseillers municipaux, relèvent du pacte de gouvernance plutôt que du règlement intérieur.

La commission des lois du Sénat a réécrit les dispositions du projet de loi relatives au pacte de gouvernance en vue d'en faire un rendez-vous en début de mandature, lors duquel les nouvelles équipes définiront les principaux fondements des relations entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres. Outre les considérations liées au fonctionnement des instances politiques et à la mutualisation des services, déjà traités, prévoir que le pacte de gouvernance traite des moyens de renforcer les solidarités financières consoliderait la portée et la cohérence de cette étape initiale. L'exercice de définition des objectifs d'un éventuel pacte financier et fiscal amène en effet les élus à prendre la mesure de la situation budgétaire et financière au sein du couple communes-communautés, et à définir la trajectoire des moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du projet de territoire intercommunal et à l'exercice des compétences par les communes et l'EPCI à fiscalité propre. Ce temps trouvera donc toute sa place dans le cadre du pacte de gouvernance en début de mandature, pour faciliter le travail des élus municipaux et communautaires dans le cadre de leur intercommunalité.

Dans la version du texte issue des travaux de la commission des lois, il est prévu que ce pacte détermine notamment les modalités de mutualisation de services, les conditions de création ou de gestion d'équipements et de services, les conditions d'engagement de certaines dépenses d'entretien, etc. Toutefois, il n'est pas prévu que le pacte de gouvernance traite d'un sujet clé du modèle intercommunal : le renforcement des solidarités financières entre les différentes collectivités. Cette composante est pourtant un élément déterminant de l'esprit communautaire, dans lequel il est important d'impliquer l'ensemble des maires. Si l'objectif partagé du pacte de gouvernance est de mieux coordonner les interventions des communes au sein de l'EPCI et de rationaliser l'organisation, la question de la péréquation financière intercommunale ne peut être éludée dans ce cadre. C'est pourquoi cet amendement, en toute simplicité, tend à garantir que le pacte de gouvernance traite des moyens de renforcer les solidarités financières dans les EPCI. La parole

territoire. Le pacte de gouvernance vise à poser en début de mandat les bases des relations entre l'intercommunalité et les communes. La commission a utilement souhaité préciser les sujets à débattre au sein du pacte de gouvernance. Comme mes collègues, je pense qu'il est important qu'à

à la prise de décision- un mot que nous n'avons pas encore beaucoup entendu ce soir. Nous sommes en train de définir le pacte de gouvernance. Il s'agit de préciser les grands principes de fonctionnement entre les communes et l'EPCI, donc

des différentes instances de cette concertation, sans rien ôter aux élus. Mme le rapporteur m'a proposé une autre rédaction, mais, avant de l'envisager, je souhaiterais entendre l'avis de M. le ministre. Quel sommes. Quel est l'avis de la commission ?

De quoi est-il question ? Si je ne m'abuse, le Président de la République a demandé au Gouvernement de désigner par tirage au sort un certain nombre de citoyens

qui pourront acquérir une valeur législative si le Gouvernement les transmet au Parlement.

Je vous remercie

quand on parle des citoyens. Je vous rappelle les termes de l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

d'aborder la relation entre les citoyens et la démocratie locale. Ce que nous souhaitons, c'est que la machine communale et intercommunale fonctionne mieux. Quand on nous renvoie à une espèce de sens naturel et inné

Le débat que nous avons en ce moment est celui qui oppose démocratie représentative et démocratie participative.

c'est une source de rajeunissement, peut-être même un bain de jouvence. Enfin, comme dans l'ancien monde, un bon vieux débat entre la gauche et la droite

avons tous oublié, moi le premier, au moment où nous nous enflammions dans ce débat essentiel, que ce pacte de gouvernance, malgré un nom qui annonce une ambition considérable, était un document facultatif Aucune intercommunalité n'est et ne sera jamais obligée de conclure un pacte de gouvernance, Dieu merci d'ailleurs ! Il est heureux que le législateur, dans sa sagesse, ait tout de même défini ce que pourrait contenir un pacte de gouvernance. Sinon, nos

on va cesser de rendre ce conseil de développement obligatoire. Cela pourrait même contribuer à faire des économies, parce que, dans la pratique, une intercommunalité de 20 000 habitants peut très bien réussir, sans conseil de développement, à associer les forces vives du territoire à son fonctionnement.

Monsieur le ministre, bienvenue dans le nouveau monde ! Le 8 septembre 2019,

de mettre un peu d'huile dans les rouages de cette loi sur le cumul des mandats et de faire en sorte que l'articulation nécessaire et indispensable entre le travail d'élu local et celui de parlementaire se joue plus simplement à travers les conseils

à la composition du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale, notamment les conditions relatives à la représentation des différentes parties du territoire, ainsi que des dispositions permettant de tendre vers la parité.

M. Arnaud de Belenet. L'alinéa 13 de l'article 1 prévoit la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de déléguer aux communes la création et la gestion de certains équipements ou services.

nous préférerons la rédaction initiale de l'article 1, qui était circonscrite à deux champs de compétence : la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

liberté » et « sur mesure ». Or l'amendement n° 442 tend à supprimer la possibilité pour les EPCI de déléguer leurs compétences à leurs communes membres dans le cadre du pacte de gouvernance.

Il doit exprimer une vision de l'EPCI sur les enjeux du territoire et développer la stratégie mise en oeuvre pour y répondre. L'objectif est double : d'une part, mobiliser l'EPCI autour d'une vision stratégique qui crée du sens pour l'ensemble des communes, donc susciter l'adhésion à un projet commun d'autre part, obtenir des engagements fermes de l'EPCI et travailler sur une stratégie qui puisse aboutir à une logique de veille sur sa bonne exécution. Quel est l'avis de la commission ?

est à M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à réintroduire dans le texte la disposition selon laquelle le pacte de gouvernance peut prévoir la création de conférences territoriales des maires sur un périmètre infracommunautaire. Ces réunions infracommunautaires auraient lieu au moins une fois par an, pour permettre un véritable débat sur les enjeux de territoire, ce que ne permet pas toujours le conseil communautaire, la détermination d'enjeux de territoire et d'objectifs à atteindre par l'EPCI et la consultation des maires sur certaines politiques de l'EPCI.

des maires, instances distinctes du conseil des maires qui permettent à certaines des communes membres d'un même EPCI rencontrant des difficultés communes de travailler ensemble et d'être consultées lorsque l'EPCI veut mettre en oeuvre des politiques les concernant. Il nous paraît normal d'intégrer ces conférences territoriales aux options du pacte de gouvernance, puisqu'elles existent déjà dans de nombreux EPCI qu'elles sont un outil utile au bon fonctionnement des intercommunalités et au respect des différences des communes qui composent celles-ci. Elles permettent également le rapprochement et le dialogue entre des communes partageant des caractéristiques communes. Il existe, par exemple, au sein de la métropole de Lyon, neuf conférences territoriales des maires, qui réunissent les maires d'une partie du territoire, à côté de la conférence métropolitaine des maires, qui réunit, elle, l'ensemble des maires des communes membres.